Cela présente le risque d'affaiblir l'indépendance de l'Ademe et de remettre en cause les liens privilégiés que celle-ci entretient avec les collectivités territoriales.

cette modification de gouvernance de l'Ademe, établissement public crucial pour la protection de l'environnement, nous paraît relativement floue. En effet, cette agence bénéficie de la tutelle des ministères chargés de la recherche et de l'innovation, de la transition écologique et solidaire et de l'enseignement supérieur.

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l'article 45 du projet de loi pour ce qui concerne la qualité de délégué territorial de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Les finalités de la loi n'exigent pas de conférer au représentant de l'État un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des activités des directions régionales ni de contrevenir aux règles d'attribution des aides de l'Ademe fixées par le conseil d'administration Cet amendement tend à garantir que cette mission confiée au préfet relève bien des compétences de celui-ci en tant que représentant de l'État et ne mette pas en péril le pouvoir hiérarchique de l'agence sur ses propres salariés, en mentionnant explicitement son rôle nécessaire de coordination de l'action de l'État et de ses opérateurs.

attribuer au préfet la qualité de délégué territorial de l'Ademe permettra, selon nous, de renforcer la cohérence de l'action de l'État en matière de transition écologique à l'échelle de la région.

demande de retrait et, à défaut, avis défavorable. L'amendement n° 554 tend à préciser le rôle de coordination du préfet de région en tant que délégué territorial de l'Ademe

vise à préciser la portée des attributions du délégué territorial de l'Ademe. En tant que délégué territorial de l'Ademe, le préfet de région aura un véritable rôle de mise en cohérence de l'action territoriale de l'agence d'une part, les objectifs qui lui sont assignés à l'échelon national et, plus globalement, les orientations gouvernementales et, d'autre part, l'activité des services de l'État dans l'ensemble des champs d'intervention de l'opérateur. Ce sera en particulier le cas avec deux politiques publiques majeures de la transition énergétique et écologique : le soutien à la chaleur renouvelable et la prévention et la gestion des déchets.

outre, il travaille déjà en bonne relation et collaboration avec les services déconcentrés de l'État et avec les préfets, dans le cadre de la mission interministérielle de l'eau et de la nature. Cette collaboration est formalisée dans un document de cadrage,

et d'une reprise en main par l'État qui ne dit pas son nom. Les modifications apportées par nos rapporteurs, tout à fait cosmétiques, n'ont pas modifié cet état de fait. Nous souscrivons au point de vue des élus membres du Conseil national d'évaluation des normes, qui ont critiqué cette disposition, la jugeant contraire aux ambitions affichées par le Gouvernement en matière de proximité et d'efficacité de l'action publique. Nous proposons donc sa suppression.

ne sont pas de nature à modifier la proposition du Gouvernement, alors, en effet, il y a un véritable problème. Si vous mettez sur le même pied le préfet de région et le préfet de département,

essayé de répondre aux problématiques soulevées par le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), en remettant le comité de bassin au centre des enjeux et en rapprochant

les projets de l'État dans la perspective de la meilleure coordination possible entre l'action des services déconcentrés et celle des agences au service des politiques de l'eau et de la biodiversité. Les conseils d'administration des agences de l'eau,

normal que les agences de l'eau tiennent compte des politiques publiques que l'État entend mettre en place. Par ailleurs, dans un objectif de meilleure coordination entre les services déconcentrés de l'État et les agences de l'eau, mais aussi d'une plus grande déconcentration, il est proposé que le préfet coordonnateur de bassin préside le conseil d'administration des agences. En fait, nous régularisons ce qui existe déjà, en pratique, depuis 2021. en pratique, depuis 2021. Auparavant, trois des six présidents étaient des inspecteurs du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). Nous ne changeons rien

territoires. Nous réaffirmons donc avec force et clarté, sur cette question des agences de l'eau, comme sur la question de l'Ademe et sur les autres points que nous verrons dans quelques instants et qui ont tous trait à l'organisation de l'État territorial et à ces mesures de déconcentration,

aux différents usages dans chaque bassin n'intègre pas explicitement la société civile, incarnée par les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (Ceser). En effet, les Ceser apportent une vision équilibrée, fruit de dialogues démocratiques sur les enjeux liés à la gestion de ces milieux. C'est pourquoi cet amendement vise à intégrer les présidents de Ceser dans les comités de bassin à partir de leur prochain renouvellement et dans les comités régionaux de la biodiversité pour renforcer l'expression de la société civile

entre des membres de la société civile organisée indépendants des pouvoirs politiques en place. Ce point est fondamental. En suggérant que les membres des Ceser soient désormais nommés par le conseil régional nouvellement élu, l'amendement adopté en commission suscite est l'indépendance politique, institutionnelle et organisationnelle du Ceser ? Quelle sera la valeur ajoutée en termes de relations de travail entre les deux assemblées, alors que la récente réforme du Conseil national a acté la suppression des quarante sièges de personnalités qualifiées, afin notamment d'assurer son indépendance et que s'exprime une attente forte en termes de démocratie participative ? Le Sénat va devoir rassurer sur ce point. ? Je veux déjà dire à notre collègue Dominique Théophile que nous sommes revenus sur le sujet de la nomination des membres du Ceser par les conseils régionaux. Son argument a donc trouvé une suite favorable dans les positions qui ont été prises lors du débat et

plutôt assidus. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été réécrite.

par décret, notamment en matière d'exigences environnementales, lorsque le législateur a confié au pouvoir réglementaire national l'application de dispositions législatives. Autrement dit, le préfet a le pouvoir d'intervenir, cadre de ce dispositif, pour déroger dans le domaine de compétences des collectivités territoriales, et non précisément dans celui de l'État. D'une part, ce renforcement des pouvoirs du préfet altère le rapport à la légalité par la création de dispositifs permettant de neutraliser la volonté du législateur, sous couvert d'adaptation locale et de différenciation, alors même que le législateur peut directement, dans la loi, prévoir ou non de renvoyer des dispositions au pouvoir réglementaire local ou national. D'autre part, renforcer la déconcentration n'implique pas, à nos yeux, de renforcer les pouvoirs du préfet. Il faut, au contraire, travailler à une reconquête de la présence de l'État dans nos territoires, dans la diversité de ses services publics, y compris par ses services déconcentrés. À nos yeux,

Le présent amendement vise à supprimer l'article 46, adopté par la commission. En effet, cet article étend le pouvoir de dérogation du préfet, reconnu par le décret du 8 avril 2020, aux normes réglementaires applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Quand bien même les matières dans lesquelles cette dérogation pourrait intervenir seraient limitativement énumérées par décret en Conseil d'État, une telle évolution doit être envisagée avec précaution au regard des règles constitutionnelles relatives au rôle du représentant de l'État, auquel l'article 72 de la Constitution confie, dans les collectivités territoriales de la République, « la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. En clair, le préfet ne pourrait contrôler et déroger dans le même temps. Par ailleurs, cet article donnerait la possibilité au préfet d'intervenir pour déroger non pas dans le domaine des compétences de l'État, mais dans celui des collectivités territoriales et de leurs groupements, lui aussi protégé par l'article 72. On peut également douter que cette mesure soit compatible avec l'article 37 de la Constitution, qui confie au seul Premier ministre le pouvoir réglementaire et qu'il peut seul ajuster, comme dans le décret relatif au droit de dérogation reconnu au préfet. Enfin, la maturité des collectivités territoriales et de leurs groupements plaide plutôt, ainsi que l'article 2 du projet de loi le prévoit, en faveur d'une extension du pouvoir réglementaire propre, qu'elles pourraient exprimer elles-mêmes de façon différenciée.

Mme la ministre.

? Il nous semble que cet amendement est largement satisfait par l'article 46, que nous avons ajouté en commission et qui prévoit la généralisation de l'information systématique des communes en cas d'évolution des services déconcentrés. La commission a sollicité le retrait

convient de renforcer le pouvoir des préfets à l'échelon départemental. Il y est fait référence à un rapport de la Cour des comptes de 2017, qui relève

l'investissement étant porté par les collectivités territoriales, communes et intercommunalités. Actuellement, ces subventions sont attribuées principalement par les préfets de région. Il est important que la proximité soit de mise, avec un rôle renforcé des préfets à l'échelon départemental,

Monsieur le rapporteur,

Les auteurs de cet amendement proposent qu'un représentant du département siège à la commission départementale des investissements locaux créée par cet article. Le département est le garant des équilibres territoriaux.

Cet amendement tend ainsi à améliorer la procédure d'octroi de ces dotations prévue dans le présent article à la lumière de l'expérience de la procédure d'attribution de la DETR, qui a montré que le rôle de la commission des élus, dans les faits, très limité. Le présent article prévoit que la commission départementale des investissements locaux rende un avis sur les projets auxquels le préfet entend donner une suite favorable. Si le dispositif envisagé est préférable au cadre prévu par la DETR- puisque l'avis porterait sur les dossiers sélectionnés, quel que soit leur montant -, cette « présélection » réalisée par le préfet réduit encore significativement le rôle consultatif de la commission des élus, dont les membres sont pourtant dotés de la légitimité démocratique. Par ailleurs, l'expérience montre que le préfet dispose d'une grande latitude dans le choix des projets retenus et n'est pas lié par les priorités établies par la commission des élus. Il peut même ne retenir aucun dossier entrant dans une catégorie inscrite dans le règlement à la demande de la commission ou qu'elle jugerait particulièrement prioritaire.

le préfet doit respecter les opérations prioritaires identifiées par la commission dans le cadre de la détermination de la programmation ; le préfet doit rendre compte à la commission de ses choix et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subvention

tandis que celles dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants ne le sont que si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen de toutes les communes de même catégorie. Lors du projet de loi de finances

et la région, avec les fonds européens. La DETR doit devenir le levier d'investissement indispensable pour les communes rurales. C'est pourquoi l'introduction du facteur démographique de la commune dans le calcul est une piste intéressante.

n'a pas compensé le retrait progressif de la présence de l'État. Or nos collectivités ont besoin d'une ingénierie territoriale en amont,

Cet amendement vise à permettre aux métropoles de coélaborer et coadopter le volet métropolitain des contrats de plan État-région, qui comporte un volet de cohésion interterritoriale.

modifier les statuts de l'établissement public, ses missions, la représentation des collectivités territoriales dans sa gouvernance, mais également définir les conditions de leur participation financière à cet établissement. À ce jour, le budget du Cerema provient, pour l'essentiel, de la subvention pour charges de service public versée par l'État, dont la baisse est sensible depuis quelques années. Une telle diminution n'étant pas compensée par les prestations payantes assurées par l'établissement public pour compte de tiers, un changement de modèle devient nécessaire pour assurer la survie de l'établissement et y maintenir l'ingénierie qui y subsiste après les réformes de ces dernières années. Deux missions d'inspection successives ont été diligentées, en 2018 et 2021, la dernière à la demande conjointe de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la cohésion des territoires, afin d'accompagner la réflexion et de préparer des scénarios d'évolution. Le premier rapport n'a pas été rendu public. Le second est en voie d'achèvement. En proposant de modifier les conditions de participation des collectivités territoriales au financement du Cerema, sans donner à voir les pistes de réflexion et les propositions issues de ces rapports, le Gouvernement n'associe pas les parlementaires à l'analyse des scénarios et des impacts financiers des mesures qui leur seront soumises, prenant le risque de faire supporter aux collectivités une charge supérieure à leurs capacités financières. La viabilité du futur modèle du Cerema reposant sur l'acceptabilité du financement par les collectivités, il paraît nécessaire d'en débattre et de légiférer en disposant des éléments d'analyse requis. Quel

acteurs territoriaux. En effet, si la participation et la meilleure intégration des collectivités territoriales sont des éléments positifs, il ne faudrait pas que le Cerema ne puisse plus répondre aux commandes des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, des agences d'urbanisme, voire de la CNR. Une telle mesure permettra au Cerema de dégager des recettes supplémentaires.

d'un amendement d'appel. Le projet de loi initial habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier le statut du Cerema et prévoir les conditions de la participation des collectivités territoriales au financement de ses missions. Le Gouvernement envisageait ainsi de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de faire appel aux capacités d'expertise du Cerema dans le cadre de la quasi-régie conjointe prévue par le code de la commande publique.

Nous défendons tous les ans, dans le cadre du projet de loi de finances, des amendements pour maintenir le plafond d'emploi de ces opérateurs à qui, par ailleurs, on attribue de plus en plus de missions. à titre d'exemple, le ministère de l'écologie a perdu plus de 4 000 équivalents temps plein depuis 2018 ; sont notamment concernés l'OFB, les agences de l'eau, Météo-France, l'IGN ou encore le Cerema. C'est pourquoi il semble indispensable qu'un renforcement des missions d'un opérateur s'accompagne de moyens humains et financiers adaptés.

d'autre but que l'affichage politique. L'article 49 en fait partie. Il a pour objet le label France Services, créé par la circulaire du Premier ministre du 1 juillet 2019, qui constitue pour l'essentiel un recyclage des maisons de services au public financées très majoritairement par les collectivités territoriales. Sous prétexte d'actualisation législative, cet article ne fait en réalité que mettre en musique l'opération d'appropriation par le Gouvernement des actions conduites par les collectivités en matière d'accès aux services publics.

que ces maisons France Services soient le retour tant attendu par les populations des services publics comme acteurs de cohésion sociale et incarnation de l'égalité républicaine dans l'ensemble de nos territoires.

dans les territoires frontaliers implique parfois des démarches administratives de l'autre côté de la frontière, qu'il s'agisse d'emploi, de prestations sociales, de fiscalité, d'études ou de formation. Prenons exemple sur différentes structures existantes qui conseillent les usagers quant à leurs démarches de part et d'autre de la frontière- je pense en particulier à la Maison ouverte des services pour l'Allemagne, à Forbach. Les bureaux France Services présents dans les territoires doivent pouvoir apporter un appui précis et concret aux administrés dans l'accomplissement de leurs formalités administratives concernant les services relevant d'autorités ou d'administrations de l'État voisin.

Aujourd'hui, dans les territoires ruraux en particulier, les intercommunalités sont extrêmement grandes, non en nombre d'habitants mais en superficie et en nombre de communes. Il me semble qu'il serait important

La création et la gestion des maisons de services au public relèvent de la compétence des communautés de communes et des communautés d'agglomération, mais cette compétence est seulement de nature facultative. Il est néanmoins aisé d'observer que beaucoup de services au public intégrés à ce dispositif sont de la compétence des communes.

savoirs, grâce à la mobilisation de l'expertise du réseau des agents, mais aussi à une meilleure prise en compte des difficultés réelles de chaque territoire. Cet amendement vise à ce que les maires soient associés en amont à tout projet de convention que signerait l'EPCI

monsieur le président.

Cela se décide sur le territoire, entre les élus et le préfet. La géographie des France Services est donc négociée localement.

Et sachez que nous sommes là pour répondre à vos besoins dans les territoires.

pour les collectivités en matière de frais de fonctionnement. L'enveloppe de 30 000 euros est largement insuffisante pour payer les salaires des personnes nécessaires au fonctionnement de la structure. Cet article a une portée normative relativement limitée. C'est la raison pour laquelle nous proposons que les usagers puissent avoir accès aux services publics proposés en moins de trente minutes, depuis leur domicile ou leur lieu de travail, en transports collectifs ou individuels.

à cette offre minimale de service doit être spécifié dans le texte que nous examinons.

Cet amendement vise à affirmer la prise en compte de trois objectifs prioritaires au niveau de la loi : la proximité géographique des usagers, l'accès aux personnes en situation de handicap et la lutte contre l'illectronisme.

la confidentialité des procédures ainsi qu'une aide réelle à remplir des dossiers dématérialisés doivent impérativement être prises en compte dans la labellisation de ces structures. Quel

à M. Dominique Théophile. Le présent amendement vise tout d'abord à rétablir la mention du référentiel France Services approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales dans l'article 27 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En effet, la notion de référentiel doit être maintenue en ce qu'elle permet d'assurer un socle homogène d'offre et de qualité de services pour chaque France Services. Le contenu du référentiel sera défini par un décret en Conseil d'État.

d'un forfait annuel de fonctionnement de 30 000 euros. L'État prend également en charge la formation des agents, l'animation du réseau ainsi que le déploiement des outils informatiques par le biais de la Banque des territoires de la Caisse des dépôts et consignations. Une attention particulière est portée aux territoires situés dans des zones de revitalisation rurale et dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. deux appels à manifestation d'intérêt ont été lancés à l'été et en octobre 2020 pour mettre en circulation quatre-vingts espaces France Services itinérants dans les quartiers de la politique de la ville et dans les zones rurales. Soumis aux mêmes critères de labellisation qu'une structure fixe, ils bénéficient ensuite d'une aide au fonctionnement identique de 30 000 euros. Enfin, l'amendement vise à abroger la restauration de l'obligation faite aux France Services de tenir compte de la situation des travailleurs saisonniers

Il s'agit de tirer les conséquences de la crise sanitaire et d'éviter aux maires de devoir contourner la loi afin de prendre part à des groupements de commandes de masques à destination de leurs agents.

commission ? Ces amendements visent à autoriser le conseil municipal à déléguer au maire la signature d'un groupement de commandes. L'idée est très intéressante, mais elle

La commission des lois a introduit la possibilité, pour l'assemblée délibérante, de restreindre la délégation consentie en matière d'admission en non-valeur à certaines catégories de recettes ou à un seuil défini par décret. Or la rédaction initiale de l'article ne faisait pas interdiction à l'organe délibérant de restreindre le champ de la délégation qu'il consent à l'exécutif local tant que le montant des admissions en non-valeur visées par la mesure reste inférieur au seuil fixé par le décret. De plus, la notion de « catégories » de titre de recettes risque de se révéler dépourvue d'application pratique. La démarche promue au niveau local vise plus simplement à adapter le périmètre au regard des enjeux financiers. S'il est possible d'envisager d'autres paramètres pour définir le champ de la délégation, cela n'est donc pas souhaitable. Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites pour retenir la rédaction initiale, qui permet de proportionner le champ de la délégation aux enjeux financiers associés.

Il s'agit d'une forme de participation nouvelle, à côté des élections des représentants, qu'il convient d'encourager. En associant chaque année les citoyens à la décision publique et en allouant une partie

à disposition des collectivités, afin qu'elles soient pleinement en mesure de vérifier le bon usage des fonds alloués.

il me semble qu'une telle disposition n'est pas forcément nécessaire, compte tenu des incidences ou des effets collatéraux qu'elle pourrait avoir. En effet, en amont, les collectivités peuvent définir un certain nombre de critères auxquels sont soumis

Cet amendement tend à élargir le périmètre des personnes morales auxquelles les collectivités peuvent céder des biens à titre gratuit. Bon nombre de ces dernières mènent des opérations de coopération décentralisée avec d'autres collectivités, mais aussi, notamment pour ce qui concerne les départements ou les régions,

pour compléter leur action extérieure. L'État peut, par ailleurs, conclure une convention internationale avec un État étranger afin d'autoriser ce type de cession. Je retire l'amendement

M. Didier Marie. Les conseils municipaux, départementaux et régionaux peuvent déléguer au maire ou au président la décision d'aliéner de gré à gré des biens mobiliers, c'est-à-dire de céder une partie de ces biens, notamment lorsqu'ils ne lui sont plus utiles ou obsolètes. Les textes en vigueur autorisent cette délégation au maire pour les biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 euros. Cet amendement vise à ne pas fixer ce montant dans la loi et à laisser aux organes délibérants le soin de déterminer la somme maximale des biens qui peuvent faire l'objet de la délégation au maire.

Le transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires au président de l'intercommunalité est possible dès lors que ces pouvoirs correspondent aux compétences transférées à l'intercommunalité. Dans six domaines, il existe un mécanisme complexe de transfert automatique, sauf opposition exprimée par tout ou partie des maires concernant leurs communes respectives, avec possibilité pour le président d'y renoncer dès lors qu'au moins un maire a exprimé son opposition. Ces choix doivent intervenir à la suite de l'élection du président de l'intercommunalité : les maires disposent de six mois à compter de cette date pour formuler leur éventuelle opposition. Une fois échus les délais initialement prévus, il n'est pas possible pour les maires ou le président de revenir sur leurs choix durant toute la durée du mandat du président. À aucun moment, le pouvoir de police administrative générale des maires n'est concerné. L'expérience des réinstallations consécutives aux élections municipales et communautaires de 2014 puis de 2020 montre que le dispositif a souvent été mal compris, en ce qui concerne tant les possibilités d'opposition que l'intérêt à ce qu'un président d'intercommunalité exerce des attributions de police spéciale pour faciliter l'exercice des compétences intercommunales- par exemple, en matière de collecte des déchets, grâce à l'adoption d'un unique règlement de collecte. Le présent amendement vise ainsi à prévoir l'organisation d'un débat au sein de la conférence des maires ou, à défaut, du bureau communautaire, en amont des décisions individuelles prises par les maires pour faire obstacle au transfert des pouvoirs de police spéciale. L'objectif est que ces choix soient préparés en bonne connaissance de cause grâce à un échange entre les élus portant sur plusieurs points : l'opportunité du transfert au président pour la durée de son mandat, eu égard aux contours des attributions de police concernées et au lien avec les compétences exercées par l'intercommunalité ; les modalités d'exercice de ces pouvoirs de police administrative spéciale par les maires ou le président d'intercommunalité, selon les choix qui seront faits, en cohérence avec l'exercice par l'intercommunalité de ses compétences. Ce dispositif ne met pas en cause les choix effectués lors des réinstallations qui ont suivi les élections de 2020. Ce débat a vocation à s'appliquer à partir des prochaines élections des

de collecte. Le présent amendement vise ainsi à prévoir l'organisation d'un débat au sein de la conférence des maires ou, à défaut, du bureau communautaire, en amont des décisions individuelles prises par les maires pour faire obstacle au transfert des pouvoirs de police spéciale. L'objectif est que ces choix soient préparés en bonne connaissance de cause grâce à un échange entre les élus portant sur plusieurs points : l'opportunité du transfert au président pour la durée de son mandat, eu égard aux contours des attributions de police concernées et au lien avec les compétences exercées par l'intercommunalité, et, d'autre part, sur les modalités d'exercice de ces pouvoirs de police administrative spéciale par les maires ou le président d'intercommunalité, selon les choix qui seront faits, en cohérence avec l'exercice de ses compétences par l'intercommunalité. Ces dispositions ne s'appliqueraient bien évidemment qu'au lendemain des prochaines élections des présidents d'intercommunalité.

présenter l'amendement n° 214 rectifié. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les agents d'un service commun constitué entre une intercommunalité et au moins l'une de ses communes membres sont placés sous l'autorité fonctionnelle de l'exécutif de la collectivité gestionnaire, quelles que soient leurs tâches. Ainsi, les agents d'un service commun porté par une intercommunalité doivent recevoir leurs instructions du président de l'intercommunalité, y compris lorsqu'ils réalisent certaines de leurs missions pour le compte des communes membres. Ce changement, intervenu en 2015, est de nature à créer des difficultés dans la mise en oeuvre des services communs, car, lorsque l'intercommunalité en est la gestionnaire, les maires des communes utilisatrices n'ont plus la garantie de transmettre leurs demandes et leurs instructions directement aux agents, même si ces derniers oeuvrent au service de leurs communes- et inversement. Le fonctionnement et la dynamique des services communs s'en trouvent fragilisés dans la mesure où leur déploiement repose sur le volontariat local et le lien avec les communes utilisatrices. Le présent amendement vise ainsi à réintroduire la précédente rédaction de cet alinéa, qui prévoyait que les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire

Je prends un exemple vécu. Une commune délègue la compétence voirie à la communauté de communes. Dans ce cas, les choses sont claires : la communauté de communes